par les élus locaux, de leur mandat a consolidé le droit à la suspension du contrat de travail des salariés qui interrompent leur carrière professionnelle pour se consacrer à leur mandat, en étendant à deux mandats la durée du bénéfice du droit à la réintégration dans leur entreprise. Toutefois, seuls les maires, d'une part, et les adjoints au maire des communes d'au moins 10 000 habitants, d'autre part, ont accès à la mesure. Cette situation contribue au déficit d'attractivité des mandats pour les jeunes et les actifs du secteur privé, et ce, particulièrement, dans les plus petites communes. Nous proposons donc d'ouvrir le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration à tous les adjoints au maire, sans seuil de population. Nous proposons également d'ouvrir ce dispositif aux conseillers départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, ainsi qu'aux présidents et vice-présidents des EPCI de plus de 10 000 habitants.

la commission ? Sur l'initiative de notre collègue Éric Kerrouche, la commission a étendu le droit de suspendre son contrat de travail à l'ensemble des adjoints au maire, indépendamment de la taille de leur commune.

pour les membres du conseil municipal, à bénéficier d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants, de personnes handicapées ou de personnes âgées.

103 est retiré. Je mets aux voix l'article 27. Conformément à l'article 44, alinéa 6, du règlement, le Gouvernement demande la priorité sur l'amendement n° 985, afin qu'il soit examiné après l'article 27. Quel est l'avis de la commission ?

Comme vous le savez, je suis moi-même particulièrement mobilisée sur le sujet. À l'occasion des débats qui se sont tenus hier soir, vous avez légitimement posé la question du traitement des indemnités de fonction dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés.

Ce minimum social, témoin de la solidarité nationale, a d'ailleurs été fortement revalorisé. Alors qu'il s'élevait à 819 euros en début de quinquennat, il a fait l'objet de deux revalorisations exceptionnelles. Le dernier décret de revalorisation, paru le 11 octobre, porte son montant à 900 euros.

S'agissant du lien entre allocation aux adultes handicapés et indemnités d'élu, comme vous le savez, ces dernières se décomposent en deux parties. La fraction représentative des frais d'emploi est destinée à couvrir les frais nécessaires à l'exercice des fonctions des élus locaux, équivalant à une forme de dédommagement. Cette partie est exclue du calcul de l'AAH, comme de celui de l'ensemble des prestations sociales, depuis l'adoption de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. quant à elle, est soumise à l'impôt sur le revenu. Elle est prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Nous avons un objectif commun : faciliter l'accès des personnes en situation de handicap, notamment des bénéficiaires de l'AAH, à des fonctions électives. Aussi nous proposons, par le présent amendement du Gouvernement, d'inscrire dans la loi le principe d'une prise en compte spécifique des indemnités de fonction des élus locaux pour le calcul de l'AAH. Il serait précisé, à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, que les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, selon des modalités fixées par décret.

par ailleurs bénéficiaires de l'AAH et ne percevant pas d'autres revenus d'activité, pourront ainsi être assurés de les cumuler intégralement avec leur allocation pendant une période de six mois.

madame la secrétaire d'État. Votre présence dans ce débat était évidemment très attendue, compte tenu de l'importance du sujet que le Gouvernement a accepté de traiter, à la demande du Sénat. effectivement d'un sujet essentiel pour faciliter la participation des personnes handicapées à la vie de la cité, par l'exercice de mandats électifs. N'ayant pas pu réunir la commission,

Mais nous souhaitons que cette mesure figure dans le projet de loi. En outre, j'avais indiqué au ministre chargé des collectivités territoriales que nous ne pourrions

tirer parti de la navette pour nous assurer que le dispositif proposé n'est pas une pure et simple transposition du dispositif déjà existant pour toute activité professionnelle reprise

pour que la commission se sente pleinement à l'aise avec la proposition que vous lui faites. Sous ces réserves, je veux vous remercier d'avoir pris à coeur cette question.

La complexité du régime indemnitaire des élus locaux est souvent relevée par ces derniers. Parmi les sujets récurrents figurent les modalités de détermination de l'enveloppe indemnitaire globale

reconnaissait : « Même si la loi n'est pas toujours d'une lecture aisée, il ne me semble pas nécessaire de tenter d'en améliorer l'écriture dès lors que l'interprétation qui est donnée est suffisamment claire et connue. Je ne vous propose donc pas de modifier la loi, mais de faire en sorte que toutes les communes soient destinataires du montant de leur enveloppe indemnitaire globale dans le mois qui suit le renouvellement du conseil municipal.

d'arrondissement, sièges du bureau centralisateur de canton, communes sinistrées, communes classées station de tourisme, communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et de cohésion sociale, communes dont la population augmente à la suite de travaux publics d'intérêt national -de majorer les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-23.

Il convient donc de préciser que la majoration, lorsqu'elle est votée par un conseil municipal, s'applique à la globalité de l'enveloppe effectivement versée au maire ainsi qu'aux adjoints et conseillers délégués, l'ensemble de ces élus étant également concernés par les caractéristiques des communes prévues par la loi justifiant la possibilité d'une majoration. La parole est à Mme Nathalie Delattre,

en les élargissant à l'ensemble des maires, quelle que soit la population de la commune, afin d'éviter tout conflit en début de mandat et en gage de reconnaissance pour le temps consacré, les frais supportés ainsi que le travail accompli quotidiennement par les maires.

Compte tenu de la remise en cause de la fonction des élus par une partie de la population, certains maires n'osent pas fixer l'indemnité maximale. Aussi la loi doit-elle fixer le montant de l'indemnité allouée au maire. Il s'agit avant tout d'éviter la polémique, mais aussi les opérations de communication purement démagogiques. L'objet du présent amendement est donc de supprimer la possibilité laissée au conseil municipal de revoir à la baisse l'indemnité de fonction du maire. Ce dernier reste évidemment libre de renoncer à une partie ou à l'entièreté de son indemnité, sans que cette question soit débattue en conseil municipal.

en effet des sujets que l'on ne peut plus expliquer à nos collègues élus, notamment les effets de seuil. La vie quotidienne du maire d'une commune de 485 habitants, qui peut avoir droit jusqu'à 600 euros

est à M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à revaloriser l'indemnité de fonction de l'ensemble des maires et adjoints des communes de moins de 100 000 habitants, et pas uniquement celle des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants.

du critère démographique dans la détermination du montant de l'indemnité n'est pas forcément pertinente, à plus forte raison quand les communes concernées ne peuvent se doter de cadres pour les accompagner dans leurs missions. Enfin, le montant de l'indemnité ne compense pas toujours la perte de salaire et le coût des charges induites par le mandat, ce qui produit un effet d'éviction de certaines catégories de la population comme les jeunes, les femmes et certains actifs, et entraîne une surreprésentation des retraités.

de monter à 80 % de l'indice 1015 l'indemnité de référence des élus. Cet amendement permet de passer à la strate immédiatement supérieure à celle qui était pour l'instant prévue dans le texte. Quel

ou 2 fois le salaire moyen, avec les responsabilités afférentes. Encore une fois, c'est une bonne chose d'opérer un correctif ce soir, mais nous restons à la périphérie de ce qu'il faudrait faire pour aller vers un véritable statut de l'élu.

de l'excellent travail qu'a fait la commission. Les intentions du Gouvernement étaient d'augmenter de 150 %, me semble-t-il, les indemnités. Bien entendu, cela de valoriser le travail extrêmement chronophage et très souvent ingrat des élus. Malgré tout, la réalité est là : si l'État peut se permettre de présenter un budget qui n'est pas à l'équilibre, ce n'est pas le cas des communes.

explication de vote. Je voudrais faire remarquer que dans les petites communes, particulièrement rurales, les maires et les adjoints au maire, en tout cas les élus, sont pour la plupart- cela a été dit cet après-midi -des travailleurs indépendants, des artisans, des personnes qui négligent parfois leur activité professionnelle pour assurer une

avec une majoration indemnitaire pour les élus locaux qui ont fait le choix d'arrêter, partiellement ou totalement, leur activité, étant donné leurs charges électives. L'indemnité de fonction versée aux maires pourrait être majorée de 40 % en cas de cessation totale d'activité et de 20 % en cas de cessation partielle, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal.

Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en oeuvre. Conformément à l'article L. 1411-5, elle est présidée par le chef de l'exécutif ou son représentant. Depuis près de trente ans, les responsabilités pour les membres de ses commissions ont été croissantes avec la montée en puissance de la décentralisation, de l'encadrement de la commande publique ainsi que le développement de politiques d'achat efficientes. Dans de nombreuses communes, la commission d'appel d'offres se réunit chaque semaine, ce qui représente une charge significativement plus importante que pour les autres commissions thématiques, et donc un frein pour les conseillers sans délégation siégeant dans cette commission. Par conséquent, il est proposé qu'un conseil municipal puisse prévoir une indemnité spécifique pour ses membres lorsqu'ils siègent à une séance de la CAO ou de la CDSP. La parole est à Mme Nathalie Delattre,

S'il s'agit d'une mesure de justice, il nous semble néanmoins que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui représentent 72 % de l'ensemble des communes françaises, nombreux sont, vous le savez, les maires qui renoncent à leur indemnité ou à une partie de celle-ci. Dans cette perspective, l'amendement que nous vous proposons vise à augmenter de manière importante la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la DPEL, appelée plus couramment « dotation élu local ». Cette dotation avait été créée par la loi du 3 février 1992. Toutefois, elle n'a été que peu revalorisée depuis lors- seulement de 10,5 millions d'euros en 2006 -, en dépit de plusieurs améliorations du régime indemnitaire des élus. La somme totale étant divisée à parts égales entre les 21 452 communes éligibles en 2019, au final la somme versée à chaque commune est de 3 030 euros, ce qui correspond à 15 % du montant maximal des indemnités annuelles. C'est pourquoi cet amendement prévoit que l'État abonde cette dotation à hauteur de 130 millions d'euros, ce qui revient à doubler son montant actuel, afin de réellement permettre aux communes d'avoir les moyens nécessaires pour financer ces est évidemment financé par le gage habituel, en souhaitant que le Gouvernement l'accepte et montre ainsi qu'il a vraiment entendu l'appel des maires de ces petites communes.

Je sais que comparaison n'est pas raison, mais, là, il en va de même. Quantité de communes n'ont pas les capacités d'augmenter l'effort en direction des élus pour relever leur indemnité. Laisser les choses en l'état

Toutefois, dans la mesure où les délibérations indemnitaires sont déjà communicables, il est proposé d'établir et de présenter l'état de l'ensemble des indemnités perçues par les élus non pas tous les ans, mais tous les deux ans, pour s'aligner sur la périodicité de la présentation du bilan social.

pour 2019- vous vous souvenez des débats perturbés par une communication inopportune sur le sujet de M. le ministre Darmanin, en plein examen budgétaire -, un rétablissement seulement partiel de la situation antérieure a pu être voté au Sénat, un système de fiscalité allégé pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Cet amendement vise à revenir sur cet entre-deux peu satisfaisant. Il s'agit de rétablir le système de fiscalité antérieur à 2017, pour ne pas pénaliser, voire punir fiscalement l'engagement fort de nos maires de France. La

est absolument intenable.

Le scrutin est clos.

à Mme Maryse Carrère. Aujourd'hui, la part écrêtée du total des rémunérations cumulées retourne au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce un mandat ou une fonction

Mme Nathalie Delattre. L'article 28 permet de moduler jusqu'à 50 % le montant des indemnités des conseillers municipaux de communes de 100 000 habitants et plus en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commissions dont ils sont membres. Cet amendement vise à étendre cette disposition à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin que cela devienne une question de principe. Quel est l'avis de

Henri Cabanel, auquel s'associe notre collègue Ronan Dantec, vise à inciter le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport portant sur la prise en compte des mandats électifs dans le cadre de la mise en oeuvre d'une réforme des retraites. Le système de retraite des élus locaux, caractérisé par l'empilement de plusieurs régimes, paraît trop complexe et peu protecteur. Il n'offre pas aux élus locaux ayant opté pour une activité professionnelle à temps partiel afin d'exercer leur mandat les contreparties suffisantes en termes de droits à la retraite. Quel est l'avis de

des élus selon leur participation. Je rappelle que cette modulation est déjà possible dans les conseils régionaux, les conseils départementaux et certaines communes, comme Paris, Lyon et Marseille. L'article 28, adopté par la commission des lois, va étendre cette possibilité aux EPCI de plus de 100 000 habitants. Néanmoins, dans un souci de clarté, nous proposons d'harmoniser la rédaction de cette disposition

Or il est un sujet que Michel Raison a abordé hier et que d'autres collègues souhaitent également voir traiter : c'est celui de l'indemnité compensatoire

Figurez-vous- vous allez vous-même être très étonné de cette évolution -que les conditions de calcul et d'attribution de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, indemnité créée dans le cadre de la politique agricole commune, sont fixées

au sein des organismes professionnels agricoles, qu'ils soient professionnels, politiques ou syndicaux, ne seraient pas prises en compte. Je traduis : un agriculteur maire

à saisir votre collègue ministre de l'agriculture, au nom de la défense des élus locaux ou de la promotion de l'engagement citoyen des agriculteurs afin que ce problème soit traité très rapidement. Bien évidemment, je veux croire qu'il s'agit d'une erreur technocratique, émanant d'une direction du ministère de la culture, et qu'aucune décision politique visant à priver les maires agriculteurs de cette indemnité compensatoire n'a été prise par le Gouvernement ! La parole est

d'accompagnement et d'aide technique engagés à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mandat. Cette possibilité est déjà ouverte en ce qui concerne les conseillers municipaux. Il nous semble normal de l'étendre aux conseillers communautaires.

Il semble naturel que cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevée sur l'enveloppe indemnitaire globale accordée, le cas échéant, au bureau, conformément aux mesures en vigueur dans les communes pour les délégations octroyées aux conseillers municipaux

pour une opération déterminée, dans l'intérêt de la collectivité territoriale. Cela peut concerner l'organisation d'une manifestation de grande ampleur, le lancement d'une nouvelle opération ou un surcroît de travail exceptionnel, en cas, par exemple, de crise ou de catastrophe naturelle. de la nature de ces mandats et de leur application sur le terrain, cet amendement vise à étendre et à élargir aux présidents d'EPCI la possibilité d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil communautaire ou métropolitain peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions. Quel est l'avis de la commission ? Favorable.

Di Folco. L'article 50 de la toute nouvelle loi de transformation de la fonction publique institue une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale, le L'organisation actuelle du CNFPT compte actuellement 29 délégations. Par conséquent, cette disposition aura pour effet d'induire la suppression de certaines délégations interdépartementales et la création de nouvelles délégations régionales. Chaque délégation est dotée d'un conseil d'orientation, composé de représentants des collectivités territoriales et des organisations syndicales des agents territoriaux. Le présent amendement a pour objet de mettre fin par anticipation aux mandats des membres des conseils qui doivent être supprimés par l'effet de la suppression des délégations concernées et de permettre la mise en place des nouveaux conseils dans les délégations nouvellement créées.

privilèges. M. le président de la commission des lois a rappelé les conditions dans lesquelles nous avons examiné un millier d'amendements. Forcément, en ayant abattu une telle quantité de travail

En effet, l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. » Or le rattachement des élus locaux au régime général et l'interprétation de la Cour de cassation assimilant les indemnités de fonction

-a rendu l'exercice d'un mandat local, même de façon partielle, incompatible avec la perception des indemnités journalières dans le cadre d'un congé de maternité. Dans les faits, les caisses primaires peuvent demander le remboursement des indemnités journalières aux élues qui ont assisté, pendant leur congé de maternité, à des

d'accompagnement psychologique. Je regrette d'ailleurs que certains responsables politiques aient raillé et moqué cette disposition dans la presse et les médias,

Comme toutes les victimes de faits d'injure ou de diffamation publiques, un élu local peut porter plainte en son nom propre et même se constituer partie civile afin de mettre en mouvement l'action publique. L'autorité judiciaire saisie de ces faits, soit le procureur de la République, soit le juge d'instruction

afin de protéger les élus locaux dans le cadre de leurs fonctions électives, y compris lorsque les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages sont relayés par le biais des réseaux sociaux. Quel est l'avis de la

L'article 30 du projet de loi prévoit, d'une part, que la commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus et, d'autre part, que la commune accorde sa protection au maire et aux élus municipaux victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Le sixième alinéa de ce même article prévoit cependant que le conseil municipal puisse s'opposer à cette protection ou en restreindre le champ pour un motif d'intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité. Cette rédaction pose deux difficultés. Premièrement, elle laisse à penser que cette possibilité de s'opposer ou de restreindre cette protection ne vise que la demande du maire et non celle des autres élus. Or on ne comprend pas très bien ce qui pourrait justifier que le maire soit placé dans une position moins protectrice que celle des autres élus. Deuxièmement, inscrire dans la loi le fait qu'un motif d'intérêt général puisse justifier une opposition ou une restriction de cette protection, et ce sans autre précision, pourrait donner lieu à un contentieux abondant en raison de la dimension politique du conseil municipal. invoqué ne sera certainement pas d'ordre financier, puisque la commune sera désormais assurée sur ce point. Il ne faudrait pas cependant que le conseil municipal retienne un motif d'intérêt général qui méconnaîtrait la présomption d'innocence ni qu'il s'érige en juge de l'opportunité des poursuites ou décide de tenir compte de l'impact médiatique de la mesure sur la commune pour restreindre la protection des élus. Dans ces conditions, il paraît plus sage de supprimer l'alinéa 6 qui pourrait donner lieu à un contentieux important. Cet alinéa est d'autant plus injustifié que la protection fonctionnelle ainsi accordée aux élus est extrêmement limitée, puisqu'elle ne recouvre que les faits de violences, de menaces ou d'outrages, et non l'hypothèse où l'élu est victime de diffamation.

ainsi libellé : La parole est à M. Alain Houpert. Les nouveaux pouvoirs confiés aux maires dans ce projet de loi qui redonne une place plus centrale à la commune ne peuvent être effectifs que si ces derniers en sont dûment informés. Cet amendement vise à mieux former les maires.

Alors que les élus se retrouvent face à des défis de plus en plus techniques dans la compréhension des politiques publiques, le système actuel est complexe et difficilement mis en oeuvre par les collectivités.

Ainsi, 70 % des répondants à la consultation réalisée par la délégation indiquent n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge des frais afférents à une formation et 99 % d'aucune compensation par la collectivité des pertes de revenus subies. Pourtant, le CGCT prévoit, dans ses articles L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12, que les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement par la collectivité, tout comme les pertes de revenus subies par les élus en raison de cette formation. L'examen des comptes administratifs des collectivités pour 2016 révèle aussi que l'effort budgétaire consacré à la formation des élus, comme le rappelle le rapport sur ce projet de loi, s'élevait en moyenne à 1,18 % du montant des indemnités de fonction- 0,83 % pour le bloc communal -, alors que le montant des dépenses de formation doit

lorsqu'un fonctionnaire exerce une activité professionnelle au cours d'une période de disponibilité, il a la possibilité de conserver ses droits à l'avancement pendant une période de cinq ans au maximum. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les droits à l'avancement d'échelon ou de grade sont conservés dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 2019. La réforme s'applique aux mises en disponibilité, ainsi qu'aux renouvellements de disponibilité à compter du 7 septembre 2018. Cependant, plusieurs catégories n'entrent pas dans le champ de la réforme, notamment les membres du Gouvernement, les parlementaires,

Cette formation comprenait un socle commun : connaissance de l'environnement institutionnel de la collectivité, connaissance des bases des missions quotidiennes- finances, budget, participation citoyenne ... -, développement personnel. Tout l'intérêt de ce parcours résidait dans un socle commun de compétences

de convertir ces droits à formation en euros. Il existe donc un risque de voir cet accès à la formation perdre en qualité, selon la valorisation monétaire de l'heure retenue pour le compte personnel de formation. Pour plus d'assurance, cet amendement garantit que le volume de formation des élus locaux soit au moins maintenu après la réforme envisagée par le Gouvernement. L'amendement n°

des élus locaux visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat est actuellement ouvert aux élus ayant une année d'exercice de mandat au minimum afin de pouvoir bénéficier de vingt heures de DIF. Or la formation s'avère particulièrement nécessaire dès les premiers mois du mandat d'un élu, surtout s'il débute dans la fonction. Par ailleurs, à la suite d'une réélection, les heures de DIF restantes doivent être utilisées dans les six mois suivant le renouvellement. Le laps de temps ainsi prévu se révèle trop court pour bénéficier d'une formation et ne permet pas de consolider la ou les formations suivies précédemment. Nous proposons d'ouvrir ce droit individuel à la formation dès le deuxième mois suivant l'élection et de prolonger sa consommation jusqu'à deux ans après le renouvellement. L'amendement L'accès au droit individuel à la formation des élus locaux est actuellement ouvert aux élus ayant une année d'exercice de mandat au minimum. Ils peuvent alors bénéficier de vingt heures de DIF et jusqu'à six mois après le renouvellement lors de l'élection suivante.

M. Jean-Marie Mizzon. Les dispositifs de formation des élus locaux seront substantiellement modifiés avec la création d'un compte personnel de formation. Pour plus d'assurance, cet amendement vise à garantir que les droits acquis au titre de l'actuel droit individuel à la formation soient maintenus au moment de la création du compte personnel de formation. Il s'agit d'une mesure d'équité pour les élus locaux, le DIF étant financé par un prélèvement sur leurs indemnités de fonction. Les deux amendements suivants sont identiques.

Améliorer la formation en lien avec leur mandat dès leur élection est d'autant plus justifié que, dans de nombreuses communes rurales, les élus exercent plus d'un mandat. Il s'agit donc d'un investissement sur le long terme. L'obligation de formation lors de la première année de mandat, prévue par le code général des collectivités territoriales, n'est pas satisfaisante, d'autant qu'elle n'est parfois pas appliquée, car limitée aux élus ayant reçu une délégation dans les communes de moins de 3 500 habitants. Selon la consultation menée par la délégation aux collectivités locales, seulement 54 % des élus ont déclaré avoir eu recours à une formation durant leur mandat. Il convient donc de prévoir, dans le cadre de l'habilitation à légiférer par ordonnance, une formation spécifique des élus lors de leur premier mandat, sans condition de taille de la collectivité locale. Toutefois, j'insiste pour que ce droit à la formation ait le moins de conséquences financières sur les collectivités locales, notamment de petite taille, et sur les indemnités des élus.

au mandat, d'une part, et de préparation à la réinsertion professionnelle, d'autre part. Il s'agit ainsi d'encourager la réinsertion des élus locaux et, donc, la fluidité de leur carrière professionnelle. L'amendement n° 670 rectifié, Jean-Marie Mizzon. Aujourd'hui, les organismes de formation, dont nombre d'associations départementales de maires, programment leurs formations en fonction des besoins locaux et des problématiques que rencontrent les élus locaux dans leurs territoires respectifs. Pour plus de clarté, l'article 31 du projet de loi prévoit la création d'un référentiel unique des formations accessibles aux élus locaux. Cet effort d'harmonisation ne doit toutefois pas conduire à exclure du marché les opérateurs locaux de formation, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. En conséquence, cet amendement vise à garantir que ce référentiel national sera adapté aux besoins des élus locaux et assurera une offre de formation accessible dans les territoires.

15 millions d'euros provisionnés, soit pratiquement 17 millions d'euros. En 2018, les seules formations budgétées par les collectivités territoriales elles-mêmes ont représenté 9,4 millions d'euros.

mes chers collègues, il est minuit passé de dix minutes. Il nous reste une cinquantaine d'amendements à examiner. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de poursuivre l'examen des articles de ce texte. Si nous restons sur le même rythme, nous devrions

par le ministère de la cohésion des territoires la mise à disposition d'une offre de formation encadrée par d'anciens élus locaux. Très souvent, les organismes de formation font appel à des universitaires ou à des experts des politiques publiques pour encadrer ces formations. Or recourir à d'anciens élus expérimentés aurait l'avantage d'assurer une meilleure reconversion et d'augmenter l'éventail de formation.

aux plans de formation mutualisés à l'échelle intercommunale, en précisant dans la loi les modalités et les modes de calcul de cette mutualisation des budgets de formation dans le cadre d'un EPCI.

à mettre en oeuvre. Malheureusement, l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Grand se limite à fixer une enveloppe de mutualisation au niveau de l'EPCI. Il ne nous semble pas, en l'état, de nature à régler les difficultés. Espérons donc que le Gouvernement pourra apporter des réponses dans le cadre de la rédaction des ordonnances. La commission demande donc le retrait

souhaitons améliorer la formation des élus locaux, qui est aujourd'hui centrale, avec notamment la complexification des politiques publiques et les difficultés d'insertion dans le marché du travail. Derrière l'objectif unique de formation, il y a bien deux chemins différents, d'une part, la professionnalisation des élus et, de l'autre, permettre à tout citoyen de s'engager dans la vie locale. Nous avons la volonté de réaffirmer que nous pouvons former les élus, en confortant leur droit à la formation, face à la technicisation de la politique, mais aussi en favorisant le retour à la vie professionnelle après la fin du mandat. Cela permet, d'un côté, d'atténuer les facteurs d'inégalités entre les citoyens et, de l'autre, de ne pas tomber dans la professionnalisation des élus, afin de renouveler la vie démocratique locale. Pour ce faire, nous proposons différentes mesures pour renforcer un droit à la formation adaptée à la fonction et à la réinsertion de tous les élus locaux. Il s'agit d'étendre la formation obligatoire dès la première année de mandat à tous les élus et non plus seulement aux élus délégués des communes de plus de 3 500 habitants de consacrer le droit individuel à la formation, à la seule formation professionnelle ; de rendre le montant consacré par les communes à la formation plus transparent, afin que cette obligation soit mieux respectée, tout en maintenant le financement du DIF par les élus eux-mêmes ; enfin, de préciser dans l'enveloppe « dotation élu local » la part consacrée à la formation et celle qui est consacrée à la revalorisation des indemnités.

en étendant cette obligation de formation. Il prévoit que la formation prévue lors de la première année de mandat soit non plus réservée aux seuls titulaires d'une délégation, mais étendue aux maires. Elle doit également pouvoir être élargie aux autres élus à leur demande. En outre, chaque assemblée locale devra définir un plan pluriannuel de formation pour la période du mandat.

ni petites communes ni grandes communes. Cet amendement concerne le principe d'égalité entre les communes, car les maires des petites communes n'ont ni agents

pour rétablir la situation antérieure et trouver une solution à ce

doit être porté dans cet hémicycle, nous attendons du Gouvernement un certain nombre d'engagements sur sa volonté de permettre aux élus locaux d'avoir une retraite digne de ce nom,

on s'interroge sur les conditions d'exercice des mandats locaux- nous avons eu de longs débats sur les indemnités des élus -, de se pencher sur les droits à la retraite des élus, en les comparant notamment avec ceux qu'ils auraient pu retirer de l'activité professionnelle qu'ils ont dû diminuer ou interrompre.

D'ailleurs, pour la personne qui perçoit soit le capital soit la rente, c'est également strictement équivalent : avec un capital placé, vous pouvez vous constituer une rente avec une rente, vous pouvez procéder à un emprunt, puisque vous aurez la capacité de le rembourser, et cet emprunt rend disponible un capital. Absolument ! Les querelles théologiques entre la rente et le capital sont donc absolument vaines ; elles ne mènent nulle part. Et tel n'est pas, d'ailleurs, le propos des auteurs de ces amendements. La commission a eu à examiner de très nombreux amendements ; un certain nombre d'entre eux ont été retirés, d'autres ont été maintenus. La difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est que le sujet n'est pas encore mûr, tout simplement parce que le Gouvernement a été saisi, à la suite de cette ordonnance dont Philippe

ce soir serait imprudent. Il vaudrait bien mieux que le Gouvernement mène une concertation pour essayer de trouver une issue à cette difficulté,

est que ces amendements soient retirés, mais au bénéfice d'un engagement du Gouvernement à traiter cette question en concertation avec les institutions concernées, qui sont dirigées par des représentants des élus locaux.

je forme un voeu, celui que les uns et les autres se parlent plus facilement. J'ai rarement vu un dossier à la fois aussi feutré

parce que je veux que chacun puisse prendre ses responsabilités. J'ai apprécié l'intervention du président de la commission des lois en lieu et place du rapporteur, mais je n'ai pas du tout été convaincu

cette possibilité de doublement du fonds retraite, alors qu'ils sentaient que le scrutin ne leur permettrait pas de retrouver leur mandat de maire. Les budgets des communes ont pu être impactés assez sévèrement, jusqu'à 12 000 euros pour une commune de moins de 100

Le présent amendement tend donc à limiter au mandat en cours la possibilité pour un élu de faire abonder son fonds retraite par la commune, afin d'éviter ce type de situations rares, mais qui ont existé, en raison de cette rétroactivité qui n'aurait pas été anticipée par les finances communales et en l'absence du regard du conseil municipal. Il faut prémunir les communes contre de tels risques budgétaires. Cette évolution devra par ailleurs s'accompagner d'une campagne d'information sur tous les droits sociaux dont disposent les élus locaux en début de mandat. Quel

Les chargés d'enseignement qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience peuvent obtenir un poste au titre de leur expérience professionnelle, comme le prévoit le code de l'éducation.

La loi du 31 mars 2015 se donne pour objectif de « faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée- sur le budget de la collectivité -au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Le législateur a paradoxalement oublié d'étendre cette obligation aux communes de moins de 3 500 habitants alors que les élus des petites communes n'ont pas les moyens des communes les plus importantes, doivent s'occuper de tous les sujets et sont en général moins rompus aux techniques administratives. La question de la formation des élus en début de mandat reste déterminante pour des raisons de fond. Il est important de créer un socle minimal autour de la prise de fonction, avec des modules que l'élu a l'obligation de suivre, visant à circonscrire le périmètre de sa fonction. En France, plus de 85 % des communes comptent moins de 2 000 habitants. Le montant prévisionnel des dépenses consacrées à la formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l'assemblée délibérante. Malgré cette évolution, on ne peut que constater une sous-utilisation des crédits destinés à la formation des élus locaux. Ce sont bien les élus des petites communes qui bénéficient le moins des crédits destinés à la formation. Face à la complexité de l'exercice du mandat à tous les niveaux face aux poids des normes, s'agissant notamment des équipements sportifs, de la performance énergétique des bâtiments, de l'accessibilité, etc. il est dorénavant indispensable que les élus qui en font la demande puissent suivre une formation dès les premiers mois d'exercice de leur mandat. Le présent amendement vise à prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement

La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative de chaque élu. Tout élu a droit à vingt heures de formation par an, cumulables tout au long du mandat. Il peut mobiliser ces heures jusqu'à six mois après la fin de son mandat. Les formations éligibles à ce titre peuvent être en lien avec l'exercice du mandat ou contribuer à la réinsertion professionnelle de l'élu local à l'issue du mandat. Si l'intérêt de ce dispositif n'est plus à démontrer, son déploiement effectif doit être soutenu à l'heure où les élus sont confrontés à une multitude de problématiques et doivent assumer des missions en nombre sans cesse croissant. En outre, les centres de formation agréés pourraient accompagner les élus dans leur reconversion dans le cadre de leur DIF non seulement pendant la durée de leur mandat, mais également dans l'année qui suit la fin de mandat. Quel est l'avis de la commission

trente premières minutes de la séance du conseil ou de l'assemblée délibérante soient réservées aux questions orales de l'opposition. Afin d'éviter des divergences d'appréciation, il est proposé de préciser la règle d'arrondi du dixième pour les demandes.

et juridiques acquises par les élus dans le cadre de leurs fonctions en leur permettant d'accéder plus facilement à une VAE, une valorisation des acquis de l'expérience. Cette reconnaissance constituera certainement un élément d'attractivité supplémentaire

Durant ce débat, les élus locaux ont interpellé le Président de la République et les membres du Gouvernement sur une pluralité de sujets, tous d'une importance cruciale pour le fonctionnement de leurs territoires et pour la vie de leurs administrés : services publics, emplois aidés, associations, réformes de la fiscalité locale et j'en passe.

avec cet amendement, nous demandons au Gouvernement de se pencher sur le sujet et, éventuellement, de donner une résonance concrète à l'invitation du Président de la République. Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement dans le cadre du grand débat national. Je sais que vous ne manquerez pas cette occasion de transformer

La préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d'eau pour la production d'eau destinée à la consommation humaine et, plus généralement, sa gestion sont des missions dont la responsabilité n'est pas clairement définie dans le droit actuel. la légitimité de l'intervention de la collectivité compétente pour l'eau potable n'est pas toujours fermement établie. Or ces missions sont essentielles pour répondre aux obligations sanitaires et environnementales auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées pour la production d'eau potable.